M. le Premier ministre. « Les Calédoniennes et les Calédoniens ont choisi de rester Français. Ils l'ont décidé librement. » C'est ce que le Président de la République a déclaré dimanche dernier. le référendum de Nouvelle-Calédonie ne marque pas la fin du chemin de pacification tracé en 1988 par Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur lors des accords de Matignon.Les Calédoniens restent divisés, malgré le passage des années.

Le premier défi est l'impératif de maintenir le dialogue avec toutes les composantes de la population, alors que les indépendantistes contestent le scrutin et refusent, pour l'heure, de reprendre langue avec le Gouvernement. Le calme impressionnant dans lequel s'est déroulée la consultation, respectée par ceux-là mêmes qui la contestaient, laisse néanmoins espérer que le fil du dialogue n'est pas rompu. Le deuxième défi est l'extraordinaire difficulté, dans la période de transition prévue jusqu'à la fin du mois de juin 2023, de construire un projet qui ne soit pas seulement institutionnel et juridique, soit de vie en commun et prenne en compte des sujets aussi cruciaux que la stratégie Nickel, l'autonomie alimentaire et énergétique, le foncier, la fiscalité et une croissance plus juste et plus soucieuse de la nature. Le troisième défi est qu'il faudra aussi répondre aux urgences des prochaines semaines, qui nécessitent un échange immédiat avec les élus calédoniens : la situation sanitaire, la situation économique, l'inquiétant déséquilibre des finances publiques. Ces défis nous sont posés dans une zone indo-pacifique devenue un enjeu géostratégique majeur, sous le regard direct d'une Chine militairement agressive, culturellement expansionniste et économiquement conquérante. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous dire comment le Gouvernement compte faire face à ces enjeux majeurs ? La parole est à M. le Premier ministre.

par le même résultat, exprimant la volonté des électrices et des électeurs de rester dans la République française. Permettez-moi de rappeler, ainsi que je l'ai dit ici même et dans d'autres instances, que je m'en réjouis.

mesdames, messieurs les sénateurs, que l'ensemble des maires, quelles que soient leurs tendances, y compris ceux qui appartiennent auxdites formations, ont organisé le scrutin. Aucun bureau de vote n'a été fermé.

sur ces travées la réserve que pouvait exprimer le Gouvernement sur le choix et la volonté qui étaient nôtres de voir la Nouvelle-Calédonie rester en France. Il n'est plus le temps de commenter tout cela.

-un projet institutionnel qui permette d'inscrire durablement, en tous les cas rapidement, la Nouvelle-Calédonie dans la République. Monsieur de quelle manière comptez-vous engager ce processus, dans un délai qui, je le crois, ne doit pas dépendre de la situation électorale actuelle- l'élection présidentielle et les élections suivantes -, tant il me paraît urgent que des signes forts puissent être envoyés à l'ensemble de nos compatriotes ?

nous avons décidé que, quel que soit le résultat du vote- par construction, nous ne le connaissions pas à ce moment-là -, l'histoire ne s'arrêterait pas, comme l'a souligné le président Malhuret. Nous avions d'ailleurs exposé toutes les conséquences et du oui et du non pour l'ensemble des acteurs et des électrices et des électeurs,

d'un contenu et d'une méthode de travail. Là encore, rien ne se fera sans dialogue. Tous les sujets sont sur la table. Nous avons fixé des échéances que vous avez rappelées, monsieur le président Buffet,

des populations et au respect des intérêts de la France, dans cette zone où, cher président Malhuret, il ne nous a pas échappé que des convoitises défavorables à notre pays sont à l'oeuvre.

La France et l'Ukraine ont une volonté partagée de renforcer leurs relations économiques, industrielles, commerciales et agricoles. C'est ce que je ressens chaque jour en tant que présidente du groupe d'amitié France-Ukraine. Cependant, l'Ukraine est un pays en guerre, dont l'intégrité territoriale est menacée depuis 2014. Tous les jours, on dénombre des morts : 13 000 depuis le conflit du Donbass, puis de la Crimée, malgré les accords de cessez-le-feu de Minsk. Sur le terrain, la situation est de plus en plus fébrile. Le groupe Wagner, à la solde du Kremlin, est sur le pied de guerre. Moscou masse des dizaines de milliers d'hommes en région frontalière, surtout des moyens militaires, en particulier des missiles de précision, qui font désormais craindre une offensive à court terme. La Russie nie pourtant tout projet d'invasion et dit procéder à des déploiements défensifs face à l'Ukraine et l'OTAN. Malgré ces dénégations, chacun sent bien que la guerre peut éclater. La diplomatie internationale est plus active que jamais. Des échanges ont eu lieu entre les chefs d'État Poutine et Biden, Macron et Zelensky, Macron et Scholz. D'autres contacts sont programmés ou en cours. L'Union européenne discute de sanctions sans précédent en cas d'attaque russe et des élus américains ont demandé hier des sanctions préventives pour dissuader la Russie d'attaquer l'Ukraine. Monsieur le ministre, alors que des bruits de bottes s'entendent aux portes de l'Europe, où en sont les négociations ? Que feront la France et l'Europe en cas de conflit ouvert ? La parole

Il faut aussi souligner la rhétorique générale alarmante de la part des autorités russes. Il faut prendre tout cela très au sérieux.

L'heure est aux échanges et aux consultations accélérées. J'ai moi-même rencontré mes collègues européens lundi à Bruxelles et mon homologue Blinken dimanche est vrai que la situation est urgente, mais il faut néanmoins garder les canaux de discussion avec la Russie pour rétablir les paramètres d'une stabilité stratégique solide en Europe. C'est la raison pour laquelle le président Macron s'est entretenu hier avec le président Poutine et qu'il doit voir en ce moment même à Bruxelles le président Zelensky. Il faut réengager des discussions substantielles sur une solution politique en Ukraine et, pour cela, retrouver le dispositif du format Normandie, la logique des accords de Minsk, celle des accords de Paris de fin décembre 2019 avant Noël, avant même d'engager des discussions politiques, prendre les mesures humanitaires qui s'imposent : à la fois la libération des prisonniers, l'ouverture de certains points de passage et la réaffirmation du cessez-le-feu. Ce serait un point important de retrait de la tension actuelle, qu'il nous est particulièrement nécessaire d'obtenir dans l'immédiat. Monsieur le ministre, face à ces démonstrations et à ces escalades, nous avons besoin d'entendre et d'avoir l'assurance que l'Ukraine est et restera la ligne rouge de l'Europe. La

Les universités doivent accueillir des étudiants toujours plus nombreux à moyens constants. Ce ciseau malthusien les fragilise et les oblige à renoncer à pourvoir des postes d'enseignant pour consacrer l'argent qui devrait être dévolu à cette masse salariale au paiement de leur fonctionnement. Ce déficit d'occupation des postes est structurel, réduit les capacités d'accompagnement pédagogique des étudiants et,, leur réussite. L'université de Nanterre aurait besoin d'un budget de fonctionnement de 25 millions d'euros, alors que sa dotation est de 11 millions d'euros. Pour ne pas renoncer à l'indispensable création d'une trentaine de postes, son conseil d'administration a voté lundi dernier, à une très large majorité, un budget en déficit de près de 3 millions d'euros. D'autres universités pourraient faire de même. Madame la ministre, je connais votre réponse : vous allez nous expliquer que jamais aucun gouvernement n'a consacré autant d'argent à l'université depuis un siècle Ma question est donc simple : comment peut-il exister un décalage aussi important entre votre perception de la situation des universités et la réalité, très difficile, vécue par les étudiants et leurs enseignants ? La parole est à Mme la ministre

je ne vais pas dire quelque chose qui ne correspond pas à la réalité ! Si le Sénat avait examiné le budget pour 2022, il se serait rendu compte qu'entre 2017 et 2022 c'est plus un milliard d'euros qui auront été bien ... Monsieur le sénateur, je ne sais pas d'où vous tenez les chiffres que vous avancez, mais je vous assure que le budget de l'université de Nanterre est bien supérieur à 11 millions d'euros : 11 millions d'euros, c'est ce que nous avons ajouté au budget de l'université de Nanterre

par tout le monde. Le Président est informé de la notification et nous continuerons à accompagner les établissements. Dernièrement, le Premier ministre et moi-même avons annoncé 100 millions d'euros supplémentaires pour soutenir les innovations pédagogiques. Nous avons récemment annoncé les lauréats du programme ExcellencES pour plus de 300 millions d'euros. Alors, oui, monsieur Ouzoulias, vous pouvez regarder les chiffres : jamais le budget de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation n'a autant augmenté que sur les cinq dernières années. Quand la situation des universités est si difficile, il n'est pas possible d'étouffer le sentiment de péril imminent par le seul déni. C'est la légitimité de la politique qui est en jeu. La véritable cause de l'abstention est là, dans ce décalage toujours plus important entre votre discours irénique et ce que vivent nos concitoyens. La parole est La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. de l'insertion. Madame la ministre, à votre arrivée au ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, vous avez eu la responsabilité du plan de relance pour l'inclusion. Après avoir mis en place un plan de soutien de 134 millions d'euros au mois d'août 2020, permettant de préserver 180 000 postes dans l'insertion et de personnes en situation de handicap au sein de 5 000 structures, 186 millions d'euros avaient été déployés pour développer les dispositifs de l'inclusion et créer de nouveaux emplois à la fin de l'année 2020. Si les résultats de cet appel à projets ont été publiés au mois de février 2021, faisant état de 3 500 projets soutenus pour 40 000 nouveaux emplois, il a été annoncé un nouvel appel à projets de 162 millions d'euros au printemps 2021. Nous attendions avec intérêt les résultats qui allaient en découler, pour pouvoir dresser un bilan global des différents volets du plan de relance pour l'inclusion. En effet, pourvoyeurs importants d'emplois et dotés d'une dimension sociale forte, les secteurs de l'insertion par l'activité économique et des entreprises adaptées permettent à de nombreuses personnes de retrouver une place dans la société. Par le travail, la formation et l'accompagnement des parcours proposés, c'est la confiance, l'assurance et la fierté retrouvée chez nos concitoyens. Ces secteurs sont aussi porteurs pour notre économie, en ce qu'ils agissent pour développer des filières de la relance, comme l'industrie, l'économie circulaire et les mobilités solidaires. Si le Gouvernement a soutenu et investi de manière inédite dans ce secteur depuis 2017 et que les objectifs semblent réalistes au vu des investissements consacrés, nous savons toutes et tous que l'exécution peut parfois être en décalage avec les engagements. J'ai pu constater que les résultats étaient au rendez-vous pour Mayotte, avec pas moins de 94 emplois créés sur le territoire. J'ai aussi vérifié les vertus de l'accompagnement de retour à l'emploi à destination de publics lors de la visite de deux structures bénéficiaires. Aussi, madame la ministre, je souhaite que vous nous présentiez les chiffres globaux du plan de relance pour l'inclusion 2020-2021 et indiquiez à la représentation nationale si les objectifs fixés seront bien atteints. La

Soilihi, dès l'été 2020, à mon arrivée au Gouvernement, nous avons mis en place le plan de relance pour l'inclusion. Il s'agissait, d'une part, de remettre à flot les entreprises de l'inclusion- 5 000 structures de l'insertion par l'activité économique et entreprises adaptées -, d'autre part, d'aider ces dernières à se moderniser, à créer des emplois et à se positionner dans le cadre de filières de relance. Ce ne sont pas moins de 500 millions d'euros que nous avons investis. À la fin de l'année 2020, nous avons recréé autant d'emplois qu'il y en avait avant la crise. D'ici à la fin de l'année prochaine, ce sont 110 000 emplois nouveaux dans l'inclusion qui auront été créés- il s'agit donc d'emplois supplémentaires. Enfin, nous sommes en bonne voie, puisque, d'ici à la fin de cette année, ce sont déjà 70 000 emplois nouveaux qui auront été créés.

En 2018 et 2019, vous proposiez que les plateformes numériques de travail adoptent des chartes facultatives- presque de bienfaisance même moment la Cour de cassation requalifiait un travailleur de chez Uber en salarié, parlant même en 2020 de phénomène d'indépendance fictive. Cette année,

concrètement des droits aux travailleurs des plateformes. Je ne referai pas en quelques minutes les débats que nous avons d'ores et déjà eus à plusieurs reprises, mais il me semble utile de préciser que le projet de directive de directive repose sur trois piliers principaux : une présomption légale et réfragable de salariat- j'y reviendrai -, une meilleure transparence de fonctionnement des algorithmes, un contrôle des effets de ces algorithmes sur les travailleurs eux-mêmes. m'interrogez sur le premier pilier. La Commission européenne a fait le choix de proposer une présomption réfragable de salariat sur la base de critères issus de certaines jurisprudences européennes. L'approche retenue par la Commission européenne pose question quant à son intérêt même pour les travailleurs, comme en témoignent mes premiers échanges avec mes homologues européens. Ces interrogations trouveront leur réponse dans le processus normal d'adoption d'une directive : c'est un temps long, qui doit permettre de nombreuses itérations entre la Commission européenne, les États membres et le Parlement européen. Toutefois, sans attendre, nous faisons le choix, en France, d'agir au plus vite pour renforcer les droits des travailleurs. Nous nous appuyons pour cela sur le dialogue social, ce qui devrait nous réunir. Je note d'ailleurs que le projet de directive s'inspire de notre modèle, en prévoyant expressément un rôle de consultation des représentants des travailleurs des plateformes.

complémentaire à notre projet de loi, qui vise à créer rapidement de nouveaux droits pour les travailleurs des plateformes. La parole Vos arguments sont spécieux, madame la ministre. Vous invoquez le dialogue social alors que votre objectif est de casser le droit du travail en imposant du précariat par la jurisprudence et par un sous-statut d'indépendance. Vous parlez de vos homologues européens, mais l'Allemagne,

Cette promesse, à laquelle je voudrais bien croire en cette période de voeux, n'est pas reflétée par la réalité à laquelle nos concitoyens sont confrontés. Par téléphone ou sur les applications informatiques, ils tentent en vain, à longueur de journée, d'obtenir un rendez-vous pour leur troisième dose. 400 000 personnes prioritaires, âgées de plus de 65 ans, n'ont toujours pas reçu cette troisième dose de rappel. Et à partir d'aujourd'hui, l'on peut aussi faire vacciner les enfants.

pourront prouver leur bonne foi afin que leur passe sanitaire ne soit pas suspendu le 15 janvier ? Sinon, envisagez-vous un report de la date prévue ?

par le ministre des solidarités et de la santé sera respectée. Vous avez raison, nous confortons le passe sanitaire, parce qu'il s'est révélé être l'un des outils importants dans la lutte contre le virus. Nous le faisons en deux temps, en ce qui concerne l'intégration de la troisième dose dans le schéma vaccinal. La première période s'ouvre aujourd'hui,

vu des moyens mobilisés pour permettre aux Français de bénéficier de cette troisième dose, je vous confirme que nous atteindrons les objectifs fixés, monsieur le sénateur.

je regrette qu'en France, pays des Lumières, on l'impose pour accéder aux bibliothèques, aux médiathèques, aux musées, quand il n'est obligatoire ni dans les transports en commun franciliens ni dans les centres commerciaux.

Le 11 juin dernier, au large des côtes corses, un crime écologique a eu lieu. Il s'agit d'un pur acte de délinquance écologique, pour reprendre les mots de vos collègues.

Elles déclaraient également : « Ceux qui ont dégazé sauvagement [ ...] sont des voyous et [ ...] seront traités comme tels. [ ...] Nous allons pouvoir agir très vite. [ ...] Vous pouvez compter sur les services de l'État pour que les enquêtes soient diligentées. Les auteurs subiront les foudres de la loi. » Nous avions fait remarquer que la zone de navigation étroite entre la Corse et la Toscane, sensible et à haut risque, car des centaines de navires s'y croisent chaque jour, était totalement dépourvue de moyens spécifiques de lutte contre la pollution, en dépit d'accidents similaires survenus par le passé. On nous avait alors promis une traque sans concession, et le Gouvernement s'était engagé à ouvrir un débat avec les élus locaux afin d'améliorer la sécurité dans cette zone. Six mois plus tard, l'urgence d'alors et la rapidité promise pour trouver les coupables font place au silence le plus total. Six mois plus tard, où en sommes-nous ? Qu'en est-il des mesures visant à améliorer la sécurité de la zone en concertation avec les élus locaux ? La

Mmes Pompili et Girardin s'étaient rendues immédiatement sur place. Un dispositif pour coordonner l'action de l'État et limiter les dégâts a été mis en place sous l'égide du préfet maritime, ce qui a permis de récupérer quinze mètres cubes de polluants en mer. mer. Une enquête a en effet été ouverte par le parquet de Marseille et confiée à la gendarmerie maritime. Les peines pour rejets volontaires sont lourdes : jusqu'à dix ans de prison et 15 millions d'euros d'amende pour l'exploitant ou le capitaine du navire. Un renforcement en matériel du centre Polmar d'Ajaccio est par ailleurs en cours, dont la dotation en équipements sera complétée à partir de 2022. Je veux saluer la mobilisation et le travail des services de l'État, en mer et sur terre, pour lutter contre la pollution maritime, et rappeler que, si notre espace maritime est l'un des plus surveillés du monde, c'est bien grâce à eux. Ce n'est

Les règles qui régissent les élections ont posé des principes afin que l'expression démocratique se fasse dans les meilleures conditions. Le législateur s'est fixé pour règle d'assurer une parfaite égalité entre les candidats. Cette règle s'applique à chacun, quels que soient sa fonction ou son statut : c'est une question de justice. Le Président de la République a le droit de convoquer la télévision. À ce droit est associé un devoir, celui de ne pas en user à des fins électorales. Combien de temps durera la mascarade qui consiste à faire du président Macron un candidat non assumé mais en pleine campagne ? Nous voyons bien que le chéquier des Français est devenu son meilleur allié, à défaut de politiques qui font sens et produisent de véritables résultats. (CSA), tatillon avec les postulants déclarés, laxiste avec l'aspirant masqué, entretient la fiction juridique ; mais gare à ne pas trop pousser l'ambiguïté ! À quatre mois de l'élection présidentielle, un candidat utilise outrageusement sa fonction de Président de la République pour obtenir une interview sur mesure, en duplex, avec des contradicteurs, sur un sujet qu'il a choisi lui-même, et diffusée le jour où sa principale concurrente devait s'exprimer sur une autre chaîne. Quelle élégance ! du vieux monde, ce privilège monarchique n'a finalement rien de nouveau ... Ne pensez-vous pas qu'il est urgent qu'un débat loyal entre tous les candidats s'installe ? Ne pensez-vous pas qu'il est urgent que le Président de la République fasse strictement la différence entre le président et le candidat, afin de parvenir à une équité démocratique attendue par nos concitoyens ?

décompté du temps de parole de l'exécutif. C'est ce qui s'est passé, comme le président du CSA le rappelait hier, lors de la dernière allocution du Président de la République. Les propos sur la pandémie ou la vaccination

Nous ne sommes pas en campagne puisque nous prenons des décisions difficiles pour le pays. Et nous allons continuer à le faire, parce que c'est là notre responsabilité Vous faites le choix de défendre le CSA. Celui-ci prendra ses responsabilités : c'est sa mission. En tout cas, l'attitude du Président de la République en ce début de campagne est révélatrice d'un président fébrile, car sa réélection est loin d'être acquise. surtout un candidat qui veut solder le débat sur son bilan, parce qu'il n'aura échappé à personne que celui-ci est désastreux, ce qui mériterait un vrai débat, et non une émission télécommandée. Si vous êtes sûrs de vous, jouez le match à fond, au lieu de tenter d'en changer les règles. La parole est à Mme Marie-Pierre Monier, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Saint-Gervais-sur-Roubion, dans la Drôme, les parents d'élèves me sollicitent, inquiets, après onze jours sans remplacement. Ce n'est là qu'un exemple d'une réalité qui concerne l'ensemble du territoire français. Dans l'Eure ou la Seine-et-Marne, les académies recourent massivement à des enseignantes et des enseignants retraités pour pallier les manques. C'est édifiant

Cette dégradation inédite des conditions de remplacement dans le premier degré s'explique facilement. C'est le prix à payer lorsqu'on poursuit des objectifs multiples- dédoublement des classes en REP et REP+, augmentation des volumes horaires de décharge -sans augmentation proportionnelle des moyens humains. Faute de créations de postes suffisantes, ces politiques, certes louables, conduisent, après avoir vidé le dispositif « Plus de maîtres que de classes », à piocher au sein des brigades de remplacement. Monsieur le ministre, qu'allez-vous faire pour résoudre ce problème ? En janvier, le travail sur la carte scolaire commencera.

pour l'école primaire en France, soit à peu près 9 % de nos effectifs. Nous les mobilisons pleinement. Contrairement à ce que vous avez dit, nous n'avons pas diminué le nombre de remplaçants en France.

le taux d'encadrement s'est amélioré, rentrée après rentrée, depuis 2017. Vous pouvez tous le vérifier, et c'est inédit dans les annales de la V République ! Tout cela se fait non pas au détriment du remplacement, mais au contraire pour le renforcer. Il est

à la fois par les facteurs structurels que j'ai mentionnés, mais aussi par des mesures spéciales, comme celles que nous avons prises en recrutant plus de contractuels l'année dernière au coeur de la crise, ou celles que nous prenons à

M. le ministre des solidarités et de la santé -ou à son remplaçant. Les projections Pasteur du 13 décembre concernant l'évolution du nombre de patients covid dans les services hospitaliers sont extrêmement préoccupantes. Les besoins en lit croissent chaque jour. Pour armer ces lits, il faut pouvoir recourir à des personnels médicaux supplémentaires. Or le contexte vous est connu : épuisement des personnels hospitaliers, urgences engorgées, hôpital proche de la saturation. Par la force des choses, les hôpitaux doivent déprogrammer des activités chirurgicales et médicales pour redéployer des personnels. Les renforts sont difficiles, pour ne pas dire même impossibles. Les médecins hospitaliers sont quant à eux contraints de prioriser les patients, avec le désarroi de devoir encore différer des soins programmés. Tout cela s'apparente à une bombe à retardement en termes de santé publique. Dans ce contexte, l'agacement des soignants croît avec leur lassitude et les questionnements éthiques ne manquent pas. Le lien de causalité n'est plus à faire entre armement de lits covid, notamment en réanimation, occupés à 70 % ou 80 % par des patients non vaccinés, et déprogrammations. Monsieur le ministre, comment comptez-vous épauler les professionnels de santé confrontés à des prises de décisions de limitation thérapeutique, autrement dénommée triage ? Le critère de vaccination peut-il être retenu comme discriminant positif

C'est parce que nous le partageons, que nous partageons ce discours de lucidité, que nous ne disons pas non plus que tout va mal. Le ministre Olivier Véran a demandé que la situation soit objectivée par une enquête sur les tensions en ressources humaines et sur le capacitaire, dont les conclusions vont être remises dans les tout prochains jours -nous vous les communiquerons. Compte tenu de cette situation, nous devons nous mobiliser collectivement, avec des réponses immédiates, d'urgence, susceptibles de produire des résultats dans les toutes prochaines semaines. D'abord, nous devons maintenir ce qui a permis aux hospitaliers de tenir jusqu'à présent, en prolongeant les majorations des heures supplémentaires et du temps de travail additionnel jusqu'en janvier 2022, ainsi que les dispositions sur le cumul emploi-retraite.

aux tensions dans les services d'urgence, en pédiatrie et dans les maternités. Le ministre a demandé aux agences régionales de santé d'être pleinement mobilisées pour accompagner les établissements en activant leurs cellules territoriales de suivi en organisant la solidarité territoriale nécessaire, notamment en mobilisant les établissements privés et les professionnels libéraux. Les actions plus structurelles, vous les connaissez,

faciliter la mise à disposition des personnels IDE des structures chirurgicales et des centres de vaccination en les remplaçant, dans ces centres, par des personnels autorisés à vacciner, mais non infirmiers

madame la ministre, sur le campus de Sciences Po Poitiers ? Les étudiants y ont dorénavant la possibilité de suivre un cours sur la sociologie de la race. Au programme : les principes du constructivisme racial, la France face à la race, ou encore la blanchité dans l'hégémonie raciale. Tout un programme Tout un programme qui, on l'aura compris, emprunte moins à Gobineau et Chamberlain qu'à l'idéologie et à la. Madame la ministre, vous dénonciez toutes ces idéologies en février dernier. Vous aviez même demandé une enquête au CNRS. enquête, le CNRS avait refusé de la mener - on peut même se demander qui décide encore dans ce pays ... Après Sciences Po Grenoble, les choix de Sciences Po Poitiers suscitent l'indignation. Et que dire de Sciences Po Paris, qui dispense trois fois plus de cours sur le genre que sur les collectivités territoriales ? On peut se demander si tel est bien le rôle de cette institution. Force est de constater que cette inversion des valeurs est désormais infusée à nos étudiants. Ma question est donc simple, madame la ministre dix mois après votre engagement à lutter contre ces idéologies, qu'avez-vous fait de concret ? Rien ! Alors que vous vous félicitez d'avoir ressuscité le débat sur ces sujets, le CNRS et Sciences Po continuent à jouer leur partition. Nous attendons des réponses, madame la ministre.

au prix de débats et de controverses, comme il est normal, car la controverse fait avancer la connaissance et l'évaluation scientifique est faite par les pairs. Mais depuis trop longtemps, nous voyons dans les établissements des événements perturbés sur le fondement de motifs partisans, idéologiques, ou de toute forme d'extrémisme. Nous voyons aussi des intitulés d'enseignement montés en épingle, au mépris du travail des enseignants-chercheurs. Nous voyons des enseignants-chercheurs et des doctorants empêchés dans leurs travaux, et ce quelle que soit leur discipline ou leur sensibilité. Et donc ? Le Sénat ne s'y est pas trompé, puisque, en octobre 2021, la mission d'information sur les influences extraeuropéennes sur la préservation des libertés académiques, présidée par Étienne Blanc, et dont le rapporteur était André Gattolin, a souligné le risque qui pesait sur les libertés académiques à cause des atteintes à l'intégrité scientifique. De la même façon,

Ma main n'a jamais tremblé, chaque fois qu'il a fallu envoyer une inspection générale, chaque fois qu'il a fallu aider des établissements à se faire évacuer. Cela faisait longtemps,

D'abord, madame la ministre, je suis heureux que nous partagions le même constat. J'espère que votre main n'a pas tremblé lorsque vous avez signé la proposition de nomination du nouveau directeur de Sciences Po, et que le ménage sera fait dans cette institution ! Ce sont tout de même les impôts des contribuables français qui financent l'enseignement supérieur, et ce sont encore les députés et les sénateurs qui choisissent les orientations budgétaires. Or nous attendons que les valeurs de la France et les Français soient enfin respectés dans ces institutions. La parole est La parole est à Mme Florence Lassarade, pour le groupe Les Républicains.

après être intervenu pour désamorcer une dispute entre voisins. Roué de coups, menacé de mort, cet élu de la République est profondément choqué. Chaque jour, en moyenne, trois ou quatre élus sont agressés. Après la mort du maire de Signes en 2019, le Sénat et l'Assemblée nationale se sont accordés sur la nécessité de mieux protéger les élus et ont adopté des mesures législatives en ce sens. Le ministère de la justice a adressé deux circulaires les invitant à recueillir avec attention les plaintes des élus et leur demandant de recourir aux sanctions prévues par la loi. Malgré ces dispositions et les instructions ministérielles, les agressions d'élus sont un phénomène en constante augmentation. En 2020, 1 276 élus ont été la cible d'agressions, soit une hausse de 200 par rapport à 2019. Force est de constater que les réponses apportées ne suffisent malheureusement pas. Ces comportements de violence ne sauraient être tolérés dans notre démocratie. Il est donc nécessaire que la justice soit plus réactive et plus sévère. Les délinquants, en particulier les mineurs, n'ont peur de rien, sachant que les condamnations sont bien souvent inexistantes. La justice est complètement embolisée, en raison du manque de moyens et du nombre croissant d'affaires à traiter Monsieur le ministre, quel signal d'autorité allez-vous envoyer ? Comment comptez-vous sanctionner les agressions d'élus ? Peut-on restaurer la crainte de la sanction ? N'est-il pas possible d'envisager, comme le propose David Lisnard, d'intercommunalité (AMF) puisse se porter partie civile lors d'agressions d'élus, afin de donner plus de poids à la procédure ? Enfin, quel dispositif d'accompagnement des élus agressés proposez-vous ?

une Europe hypocrite, qui faisait passer la raison diplomatique et économique avant la sauvegarde des peuples, de la justice et du droit. Monsieur le ministre, il serait impensable aujourd'hui que reste dans l'Histoire un camouflet

La situation est trop complexe pour la réduire à une guerre de civilisation ou de religion. C'est bien davantage un conflit ethnique et territorial. Le bloc turco-azéri menace l'existence même de l'Arménie. Le pays a besoin d'aide matérielle pour garantir la sécurité de ses frontières. Les atrocités de la guerre- exterminations, décapitations -laissent la place à une violence quotidienne au sein des populations civiles arméniennes, confirmée par le défenseur des droits d'Arménie. Les autorités de ces deux Républiques, rencontrées sur place ou au Sénat, demandent que la France prenne toute sa place dans le groupe de Minsk, afin d'aboutir à l'établissement d'une paix durable. Les coprésidents se sont réunis en novembre, et les discussions doivent maintenant aboutir à des actes. Hier, l'Arménie a déclaré vouloir nommer un émissaire pour la normalisation de ses relations avec la Turquie. Ma question est simple, monsieur le ministre. Un cessez-le-feu a été signé il y a un an sous l'égide de la Russie, sans les représentants du groupe de Minsk. Au-delà des déclarations, que fait votre gouvernement pour obtenir la libération des prisonniers et apporter un soutien matériel aux populations ?

Il est donc urgent de progresser sur les différents volets du conflit : les prisonniers, les disparus, le déminage, la préservation du patrimoine et la délimitation des frontières. Il faut essayer de trouver le chemin d'une confiance entre les deux acteurs. Nous y travaillons.

une culture commune et une solidarité particulière, qui s'est manifestée la semaine dernière lorsque le ministre délégué Jean-Baptiste Lemoyne a signé, à ma demande, une feuille de route avec les autorités arméniennes pour renforcer notre coopération dans le domaine de la santé, de la connectivité connectivité et de l'énergie, avec le soutien de l'Agence française de développement. Ainsi, la France continuera à jouer ce double rôle de responsabilité au sein du groupe de Minsk, et donc d'équilibre, et de solidarité concrète avec le peuple arménien.

Il y a des périodes dans l'histoire où il faut choisir son camp. L'an dernier, notre assemblée, en votant à l'unanimité moins une voix la demande de la reconnaissance de la République d'Artsakh, a choisi le sien, celui de la démocratie.

familles séparées pendant les fêtes de Noël : voilà ce qui attend les usagers de la SNCF après le préavis de grève déposé par certains syndicats pour ce week-end. Les méthodes de maître chanteur sont de retour, comme chaque année pendant cette période si sensible, avec des revendications diverses, confuses et corporatistes. Au moment de l'ouverture à la concurrence et des efforts notables du président Farandou et de ses équipes pour essayer de réformer l'entreprise ferroviaire historique nationale, c'est un suicide

Tout ça pour ça ! Autant d'argent public pour un seul et même résultat : l'échec dans l'amélioration de la qualité du service public ferroviaire. Ma question est toute simple, monsieur le ministre : comment le Gouvernement peut-il accepter cela ?

a fait des propositions de revalorisation des salaires, notamment des bas salaires, et proposé des primes pour lutter contre l'inflation et la sous-activité liée au covid. Un accord a d'ailleurs été signé la semaine dernière par l'UNSA et la CFDT. Vous l'avez dit également, l'État a été au rendez-vous depuis 2017, en réinvestissant plus de 75 milliards d'euros sur dix ans pour régénérer le réseau, sauver les petites lignes ferroviaires ou encore relancer les politiques du fret ferroviaire et des trains de nuit. Cette grève, monsieur le sénateur, si elle existait, elle serait incompréhensible. Elle constituerait un sacré cadeau fait à la concurrence, au moment où celle-ci arrive sur le réseau grande vitesse, et serait une mauvaise manière faite aux Français, qui, par millions, ont d'ores et déjà réservé leur billet à l'approche des fêtes de Noël. Vous le savez, monsieur le sénateur, la direction de la SNCF a fait savoir qu'elle restait à l'écoute des organisations, et je fais le pari, ici et maintenant, de la responsabilité des syndicats cheminots. La parole est à M. Monsieur le ministre, nous arrivons au même constat : vous avez mis les moyens, et ce « quoi qu'il en coûte », mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Ce qui se passe dans le ferroviaire est à l'image de ce qui se passe en France dans ce quinquennat de l'échec et du déclin. Ségur de la santé, Beauvau de la sécurité, États généraux de la justice : autant d'argent public distribué sans résultat. La situation se dégrade, le pays est en tension, les Français n'en peuvent plus

Ce rapport, dense et documenté, fait un état des lieux précis de la situation actuelle. Pour 2020, 26 000 personnes étrangères ont déposé une telle demande. Selon ce même rapport, des ressortissants issus de pas moins de 127 pays différents ont demandé à bénéficier du dispositif. Ainsi, tour à tour, on trouve des ressortissants algériens, ivoiriens, congolais, guinéens, géorgiens, maliens, comoriens, marocains, tunisiens, mais aussi émiratis, canadiens, américains, des pays où la médecine ne laisse pas Il ressort clairement de ce travail qu'une partie des demandeurs font un usage systématique de cette procédure pour obtenir un titre de séjour, notamment lorsqu'ils ont été déboutés du droit d'asile. Plus largement, ce rapport pointe du doigt une utilisation dévoyée, et même détournée, de l'accès à notre système de soins offert par la France aux étrangers. Monsieur le ministre, que répondez-vous à l'OFII, qui s'inquiète tant du coût que de la façon dont la procédure d'admission au séjour est dévoyée par une partie des demandeurs ? Surtout, quelles mesures comptez-vous prendre pour lutter véritablement contre ce détournement ?

La séance est reprise. La parole est à Mme Marie-Christine Chauvin, pour une mise au point au sujet d'un vote.

J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein des éventuelles commissions mixtes paritaires chargées d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la protection des enfants et du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation et portant habilitation du Gouvernement à compléter par ordonnance les règles organisant le dialogue social avec les plateformes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 L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants

En effet, la diversité des situations rencontrées oblige à privilégier des approches pluridisciplinaires. C'est pourquoi le référentiel de la Haute Autorité de Santé (HAS), pour pertinent qu'il soit, ne saurait s'avérer suffisant.

scientifiques liées aux procédures de la Haute Autorité de santé, toutes les garanties aussi en matière de participation, une première version de ce référentiel étant soumise au débat public et à la contribution de l'ensemble des parties prenantes. Il a été adopté et sachez, pour être totalement complet, que le futur groupement d'intérêt public, la future instance de gouvernance dont nous allons parler à l'article 13, aura pour mission parmi d'autres d'assurer la formation

Il s'agit de préciser dans la loi que les conseils départementaux seront régulièrement consultés pour l'élaboration dudit référentiel.

la commission ?

Selon l'étude d'impact du projet de loi, le recours à la collégialité doit permettre « de mettre fin à l'isolement du juge dans les dossiers en assistance éducative les plus complexes Or, laisser à la seule initiative du juge la possibilité de demander la collégialité ne permettra pas de répondre complètement à cet objectif.

Le juge des enfants, qui juge seul, ne tranche pas un litige entre des parties, mais ordonne des mesures destinées à protéger un enfant en danger. Dans cette procédure d'ordre public, son seul objectif est de prendre toute mesure nécessaire à la préservation des besoins fondamentaux de l'enfant. Contrairement à un litige commun en droit civil, le juge ne rend pas une décision définitive pour régler un différend ; il ordonne des mesures, qui sont, par nature, provisoires et évolutives selon la situation de l'enfant. Dans ce cadre, le recours à une formation collégiale présente certes un intérêt, lorsque le juge fait face à un cas particulièrement complexe, mais ce dernier doit être le seul à pouvoir l'apprécier. Confier aux parties le droit de demander une formation collégiale risquerait de cristalliser des conflits pendant la procédure et de rendre la collégialité quasi systématique. En effet, il y a de fortes chances que les parents qui ne souhaitent pas que leur enfant soit confié demandent une formation collégiale, dans l'espoir que celle-ci contredise le juge saisi de l'affaire.

en ces termes : « En matière d'assistance éducative, si la particulière complexité d'une affaire le justifie, le juge des enfants peut, à tout moment de la procédure, ordonner son renvoi à la formation collégiale du tribunal judiciaire qui statue comme juge des enfants. La formation collégiale est présidée par le juge des enfants saisi de l'affaire. » Quel est

104 décisions de justice n'étaient pas exécutées et constate que cette pratique de non-exécution n'est pas récente : elle est récurrente depuis 2016. Lorsque les décisions sont exécutées, les délais d'exécution sont parfois excessivement longs. sociales (IGAS) rendait un rapport sur les délais d'exécution des décisions de justice en matière de protection de l'enfance et faisait état d'une tendance à l'accroissement de ces délais. À titre d'exemple, s'agissant des mesures d'action éducative en milieu ouvert, un tiers

Ce retour d'information vers le juge nous semble essentiel, de même que la sensibilisation aux conséquences de délais d'exécution excessivement longs, car chaque mesure non exécutée revient à laisser un mineur en situation de danger.

Sauf que le caractère exécutoire des décisions du juge est déjà posé dans le droit civil. L'inscrire, par ces amendements, dans la loi n'apportera rien au droit positif ni à leur exécution en pratique, se heurte à la difficulté de trouver une place d'accueil pour l'enfant. Cette disposition est donc satisfaite et sans effet par rapport à l'existant. Quant à l'information du juge, elle est déjà possible. Elle est d'ailleurs largement renforcée par l'article 8, en

avec les travailleurs sociaux, n'est pas une insulte. Pour l'avoir vécu, il arrive très souvent que les mesures d'assistance éducative ou les mesures d'instruction qui sont ordonnées

L'avocat accompagne les enfants dans les procédures relatives à leur situation. Je n'y reviendrai pas dans la discussion des prochains amendements : l'avocat formé et spécialisé dans la défense des enfants permet de préparer l'enfant aux audiences, de donner une place à la parole de l'enfant ou d'exprimer ce que ce dernier n'ose pas toujours dire lors d'audiences d'une grande solennité ; il constitue enfin un repère de confiance et un repère stable, à la différence des juges, qui- ce n'est pas de leur fait ! -sont marqués par une grande rotation, la durée moyenne

Bien sûr, il peut être difficile d'avancer tout de suite dans cette direction : les moyens manquent, nombre d'avocats ne sont pas formés, les formations spécialisées se mettent tout juste en place dans les différents barreaux, mais c'est un horizon qu'il nous faudra atteindre. L'État doit envisager un grand plan de formation et d'investissement à moyen terme. C'est à lui que je C'est à lui que je m'adresse dans cette intervention liminaire. Il faut rendre possible l'accompagnement systématique des enfants par un avocat, car chaque enfant doit pouvoir être soutenu dans l'expression de sa parole et dans la défense de ses intérêts fondamentaux.

d'introduire un troisième alinéa à l'article 375-1 du code civil, afin de permettre l'audition systématique du mineur capable de discernement- nous reviendrons sur cette notion si vous le souhaitez -par le juge des enfants en assistance éducative.

Par ailleurs, cet amendement vise à introduire un quatrième alinéa modifiant le texte issu de la commission des affaires sociales du Sénat pour y ajouter, aux côtés de la désignation par le juge des enfants d'un avocat pour l'enfant capable de discernement, la désignation par ce même juge d'un administrateur pour le mineur non capable de discernement.

ou des parents. Une telle priorisation de la demande de l'aide sociale à l'enfance ne serait pas compréhensible, en outre, pour les parties à l'audience en assistance éducative. En tout état de cause, le juge des enfants fera droit à cette demande de désignation, si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant, et il devra motiver sa décision de ne pas y faire droit.

la Défenseure des enfants a précisé en 2008 que « cette notion recouvre la capacité pour l'enfant de comprendre ce qui se passe, d'appréhender la situation qu'il vit, de pouvoir exprimer ses sentiments à ce propos ». La jurisprudence l'entend comme la capacité intellectuelle à comprendre le sens

marqués par de fréquentes ruptures dans les modalités de prise en charge. Si les changements peuvent être motivés par des raisons légitimes, il arrive malheureusement qu'ils le soient par des considérations extérieures à l'intérêt supérieur de l'enfant. Or ils peuvent perturber l'enfant et susciter des ruptures de prise en charge. Aussi, nous nous félicitons que l'article 8 tende à renforcer l'information du juge en cas de changement du lieu de placement de l'enfant décidé par les services de l'aide sociale à l'enfance. Pour autant, nous souhaiterions que le juge soit consulté, et non plus seulement informé.

avant un changement de lieu de placement, sauf en cas d'urgence. Les changements de lieu de placement peuvent avoir d'importantes conséquences sur l'enfant. Il paraît normal que le juge des enfants qui suit l'enfant soit informé, mais aussi qu'il puisse donner son avis

peut avoir d'importantes conséquences sur l'enfant, même si elle est justifiée. Il apparaît donc pertinent que le juge des enfants ne soit pas seulement informé, mais « consulté », et qu'il puisse donner un avis sur le changement de lieu de placement. lieu de placement. Une telle décision est souvent prise pour protéger l'enfant. Un délai de quinze jours durant lequel le juge peut donner son avis est donc prévu afin de ne pas causer de préjudice à l'enfant. En l'absence de réponse, le changement de lieu de placement serait considéré comme approuvé. Il s'agit, vous l'aurez compris, de protéger l'intérêt supérieur de l'enfant.

Mes chers collègues, les mots ont leur importance et, en parlant de lieu « de placement », nous oublions tout le reste pour l'enfant. Au-delà d'un placement, c'est un nouveau lieu de vie pour le jeune, un lieu pour panser les plaies du passé,

peuvent être effectuées sur l'initiative de l'ASE, si celle-ci en justifie la nécessité devant le juge, mais la rédaction ne précise pas sur quel fondement cette justification devra se faire. Dans son avis, la Défenseure des droits estime qu'un renvoi à l'article 375-7 du code civil serait opportun.

en cas de changement du lieu de placement, je souhaite rappeler que les choses sont bien encadrées : lorsque l'ASE envisage de modifier le lieu de placement, la loi prévoit déjà que le service doit en informer le juge, qui

en prenant en compte le maintien des liens entre frères et soeurs, mais il ne fait pas référence à l'obligation pour l'ASE de justifier sa décision de séparation, comme le prévoit l'article 8. Raccrocher cette disposition de l'article 8 à celle du code civil n'apparaît donc pas opportun. Par conséquent, l'avis est défavorable.

dispose : « L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de 21 ans à son domicile.

sont directement employés par les départements. Il convient de garantir aux assistants familiaux une rémunération mensuelle égale au SMIC, d'instaurer une nouvelle indemnité en cas d'accueil non réalisé et de maintenir une rémunération en cas de suspension

Continuer de précariser ces professionnels n'est pas acceptable ; il est nécessaire de garantir à tous les assistants familiaux le salaire minimum de croissance mensuel. C'est pourquoi il convient de supprimer la mention

: La parole est à M. Xavier Iacovelli. Nous le savons, la mission des assistants familiaux est centrale dans la prise en charge des enfants et des jeunes sous protection. Les assistants familiaux mènent leur mission avec dévouement, parfois dans des conditions difficiles, avec des salaires plus que modestes, comme on vient de La formation des assistants familiaux est nécessaire, puisque les parcours de vie des enfants et des jeunes protégés dont ils ont la charge sont complexes et parfois chaotiques. Actuellement, dans le droit, il est prévu une formation pour les assistants maternels et un simple stage préparatoire pour les assistants familiaux. Le présent amendement vise donc à renforcer la formation des assistants familiaux en amont de l'accueil des publics ciblés, en laissant le soin au Gouvernement de fixer par décret le contenu et les modalités de validation de cette formation. Les enfants et les jeunes placés constituent un public fragile qui nécessite un accompagnement et une prise en charge efficaces. Tel est l'objet de cet amendement d'appel.

déjà satisfait : il existe déjà une formation préparant au diplôme d'État d'assistant familial, qui s'effectue après le stage préparatoire, et dont le contenu, la durée et les conditions de validation sont prévus par décret.

à préserver l'ensemble de la famille d'accueil et, par conséquent, à limiter les risques de maltraitance psychologique ou physique des enfants confiés. Il s'agirait d'offrir un temps de repos

Mis en place pour répondre à une forte attente de ces professionnels de la protection de l'enfance qui se voient confiés des enfants ou des jeunes au profil complexe, ce dispositif permet d'éviter l'essoufflement de ces assistants familiaux qui sont extrêmement sollicités et mobilisés.

Le second est lié au métier d'assistant familial. Ces professionnels sont souvent très sollicités par les services de l'aide sociale à l'enfance afin d'assurer l'accueil d'enfants au profil complexe,

C'est un temps bénéfique pour eux et pour leurs familles, qui permet d'éviter une perte de sens et, dans le pire des cas, une exaspération face à l'enfant confié. Cette proposition a donc un intérêt partagé. Surtout, elle permet une continuité et une stabilité de l'accueil de l'enfant, parce que le professionnel reste disponible et serein.

vise à insérer une phrase à l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles afin d'inscrire dans la loi la participation des assistants familiaux à l'information des équipes d'accompagnement médico-social et de l'autorité judiciaire. Les assistants familiaux sont au coeur de la vie de l'enfant qui leur est confié. Pourtant, ils n'ont souvent aucun lien avec la procédure judiciaire qui le concerne : ni en amont ni en aval. Avoir connaissance des informations figurant dans le dossier,

difficile de créer une bonne relation entre l'enfant et l'assistante familiale qui l'accueille. En aval, les assistants familiaux côtoient l'enfant tous les jours. Ils sont donc les mieux placés pour parler de leurs évolutions, de leurs récits, de leurs rapports aux autres enfants et aux adultes. Pourquoi ne sont-ils pas entendus de manière systématique pour évoquer les signes de fragilité, par exemple, ou de consolidation des enfants dont on leur confie la garde ? Il conviendrait donc, dans l'intérêt supérieur de l'enfant,

par le droit. L'article L. 421-15 du code de l'action sociale et des familles prévoit en effet une obligation de formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis.

Le Gouvernement s'est permis d'écrire en janvier 2020 à l'ensemble des présidents de conseils départementaux

concerne la base nationale d'agrément que ce texte instaure ; vous avez décidé en commission de l'étendre aux assistantes maternelles

Ainsi, un assistant maternel ou familial qui se voit retirer l'agrément ne pourrait pas, même s'il en fait la demande dans le même département ou dans un autre, se voir octroyer un nouvel agrément avant l'expiration d'un délai approprié. Les modalités de mise en oeuvre de cette disposition, s'agissant, notamment, de la durée d'opposabilité du retrait, seront définies par décret en Conseil d'État.

un an minimum. Les services du département sont contraints d'instruire la demande rapidement, sans que les conditions d'accueil des enfants aient pour autant évolué depuis le retrait ou le refus d'agrément.

des enfants en donnant aux personnes qui ont fait l'objet d'un refus ou d'un retrait d'agrément le temps nécessaire au mûrissement de leur projet ou à la

attestant de leurs capacités à assurer la santé, la sécurité, l'éveil et le développement des enfants pendant le temps d'accueil.

madame Meunier,

Bien évidemment, nous avons pris connaissance des précautions prises et des limites posées dans cet article : avis du médecin de prévention ; possibilité de prolonger cette activité à la demande de l'assistant familial prolongation uniquement pour l'accompagnement du mineur ou du jeune majeur jusqu'à ses 21 ans. Il s'agit ici d'une profession qui a ses spécificités, en particulier un lien très fort entre l'enfant et l'assistante familiale. Si nous partageons pleinement l'objectif d'éviter les ruptures d'accueil

Être assistante familiale, ce n'est pas être grand-mère ! À notre sens, cet article est une façon de gérer une nouvelle fois la pénurie : le nombre d'assistantes familiales et de familles d'accueil est insuffisant ; plutôt que de travailler sur l'attractivité de ce métier, sur un statut plus favorable, sur de vraies revalorisations salariales, vous leur proposez de travailler plus longtemps. Cet article 11 n'est d'ailleurs que la conséquence logique des articles 9 et 10, dans lesquels vous ne proposez rien pour améliorer réellement la situation professionnelle de ces femmes. Cela a même été souligné par le rapporteur

exerçant une activité professionnelle d'accueillir des enfants chez elles au titre de l'aide sociale à l'enfance. Sans exercer à proprement parler le métier d'assistante familiale, elles pourraient accueillir des enfants.

Je ne sais pas si les représentants des assistants familiaux sont les meilleurs interlocuteurs pour discuter de ce sujet. En effet, l'amendement ne vise pas tout à fait la profession d'assistant familial : ce sont des familles dont les

on n'a pas de liste des tiers dignes de confiance dans les départements. Une

Une telle mesure s'avère d'autant plus utile qu'elle permettra de s'assurer de la bonne identification des grandes priorités pluriannuelles d'action en matière de PMI, et ce en concertation avec les départements. Cependant, la commission des affaires sociales a fait le choix d'imposer comme contrainte supplémentaire que la définition de ces priorités soit nécessairement pensée conjointement par le ministre de la santé et par les départements. C'est la raison pour laquelle, par cet amendement, nous souhaitons revenir sur la remise en cause du pilotage par l'État qu'induit cette modification. Il nous semble en effet préférable de rétablir la rédaction initiale de l'article, afin de garantir une articulation efficace entre les priorités de santé publique identifiées au niveau national.

Il semble effectivement indispensable d'associer l'assurance maladie au pilotage de la politique de protection maternelle et infantile. On le sait, cette politique a non seulement souffert des désengagements financiers des gouvernements successifs, mais également des réductions de dotation des départements.

ses travaux, la commission a su trouver une rédaction qui se prémunit de toute incohérence juridique, puisque, après définition conjointe avec les départements, le ministre arrête formellement les priorités. Surtout, dans la mesure où les départements sont les acteurs principaux

prévoit que tout cela se fasse en concertation avec les départements.

de ces amendements ;

Cohen, sur l'article. Par cet article, le Gouvernement propose de regrouper les multiples instances nationales qui oeuvrent dans le champ de la protection de l'enfance. Le pilotage de la protection de l'enfance au niveau national est en effet plutôt défaillant. La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant a créé le Conseil national de la protection de l'enfance (CNPE) qui était très attendu, à l'époque, par l'ensemble des actrices et des acteurs concernés, pour améliorer la gouvernance des politiques. Le bilan, quatre ans plus tard, est plutôt décevant. Il n'y a pas vraiment d'amélioration de la situation ; on constate plutôt une certaine dégradation. L'article 13 prévoit donc de fusionner dans un groupement d'intérêt public plusieurs structures nationales, dont l'actuel Conseil national de la protection de l'enfance- j'en profite pour saluer le travail de notre ancien collègue Georges Labazée, vice-président

Si l'on souscrit à l'idée d'un pilotage national de la protection des enfants qui intègre l'ensemble des structures qui agissent dans ce domaine, se pose la question de la place des départements et de l'État dans cette compétence partagée.

à la hauteur des besoins, ce pilotage de la protection de l'enfance au niveau de l'État ou des départements ne sera pas opérationnel et ne modifiera pas la situation en profondeur. Nous ne sommes pas contre ce regroupement, à condition de dégager des moyens

de Laurence Cohen concernant cet article 13. Celui-ci s'inscrit dans la volonté de mieux piloter la politique de protection de l'enfance et

la réforme de la gouvernance nationale, dont le sens profond est de renforcer le pilotage et de nous doter, exactement comme vous l'évoquiez, monsieur Savary, d'un outil

dans les avis que je donnerai. Je me suis engagé auprès de M. Sauvadet, président de l'ADF, que je suis allé voir au lendemain de son élection en Côte-d'Or, sur le fait que le président du nouveau groupement sera un président de département.

Une coordination des services de l'État, conduite par le préfet de département, devrait permettre une plus grande cohérence et la mobilisation des différents acteurs qui concourent à la protection de l'enfance.

L'article 13 dresse toutefois une liste de personnes qui y siégeront : des députés, des sénateurs, des représentants des conseils départementaux, des représentants d'associations oeuvrant dans le champ de la protection des droits des enfants et des magistrats. Le nombre de parlementaires y était même précisé Alors que le rôle du CNPE est d'émettre des avis et de formuler des propositions relatives à la prévention et à la protection de l'enfance, il nous semble important qu'une place soit accordée aux avocats afin de faire vivre les droits des enfants.